La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur la politique du logement dans les outre-mer à la demande de la délégation sénatoriale aux outre-mer.-- Je vous rappelle que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté. Monsieur le Ministre. Si vous le jugeait nécessaire de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes. L'orateur disposera alors à son tour d'un droit de répartis pour une minute. Voilà la parole et tout d'abord aux orateurs de la délégation sénatoriale aux outre-mer qui a demandé ce débat et monsieur Stéphane Artano, président de la délégation sénatoriale aux outre-mer pour trois minutes. Monsieur Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les besoins en logement dans les outre-mer sont criants. En 2021 notre délégation consacré un rapport détaillé en écho au constat d'échec, dressé par la Cour des comptes concernant le plan logement outre-mer diplôme Face à la gravité de la crise du logement et pour contribuer à la réussite du plan de, du gouvernement. Notre délégation a procédé à un travail très approfondi de contrôle et de proposition sur cet aspect fondamental dans la vie quotidienne de nos concitoyens le fort investissement de nos collègues rapporteurs que je salue. Dans ce travail, les a conduits à élaborer un véritable programme d'action pour reconstruire cette politique. Leurs propositions sont articulés autour de 3 axes majeurs premièrement refonder les cas de rédaction de la politique logement outre-mer pour la rendre plus efficiente. assurer un habitat pour toutes les populations dans leur diversité ont enfin faire de l'habitat ultramarins un modèle d'adaptation et d'innovation capable de répondre aux nouveaux défis de la politique du logement en particulier celui du vieillissement dans certains territoires et du réchauffement climatique. Après le report de ce débat pour des raisons sanitaires liés à un an, nous nous félicitons de sa tenue car le diagnostic est toujours d'actualité. Et la volonté de nos rapporteurs de rompre radicalement avec la méthode descendante qui a prévalu au profit d'une approche territorialisée fondée sur une évaluation fine des besoins exprimés par les collectivités elles-mêmes et doté d'un pilotage permettant une meilleure coordination et concertation locale apparaît paraît toujours aussi pertinente. Je souhaiterais insister sur 4 points. Il faut d'abord diminuer le coût des opérations immobilières dans nos outre-mer notamment avec la nécessité de libérer davantage de foncier aménagé ce problème reste d'ailleurs commun à l'ensemble des territoires. Par ailleurs, le chantier de l'adaptation des normes doit être accélérée l'inadaptation normative et ton là encore un des facteurs de renchérissement des coûts, un travail important reste à conduire avec la Commission européenne nous savons le travail mené par la Nouvelle-Calédonie et de ce point de vue précurseur et pourrait servir de modèle en octobre. Vous nous aviez Monsieur le Ministre confirmez que votre objectif était de faire évoluer certaines normes européennes, où en est-on aujourd'hui. Après la présidence française de l'UE et la présidence de la conférence des RUP en 2022. Troisièmement, on doit s'atteler aussi à la résorption des habitats indignes de la République au nombre de 110.000 dans les départements d'outre- mer. Le phénomène est de plus en plus diffus. Les opérations d'auto-construction et d'auto-réhabilitation peuvent apporter des réponses et pour autant, elles sont encore trop peu utilisé, notamment du fait du manque de soutien au niveau des assurances. enfin il est nécessaire d'accélérer la construction des logements sociaux et très sociaux. Faut-il rappeler que seuls 15% des ménages des Drôme résident dans des logements sociaux, alors qu'ils sont éligibles à 80% pour les logements sociaux, et 70% pour les logements très sociaux. Le plan de fixer un objectif de 30% de logements très sociaux. Monsieur le Ministre où en sommes-nous à l'heure actuelle, quel bilan dressez-vous du plan logement outre-mer 2019 2022. Quelles initiatives avaient aux prises à la suite des rencontres avec les bailleurs sociaux et les acteurs majeurs que sont la Caisse des dépôts et Action Logement, quelles sont enfin les perspectives pour les Outre-mer en 2023. Permettez-moi d'insister sur la situation à Mayotte et en Guyane. Car le manque de logements et la multiplication des bidonvilles en d'innombrables répercussions notamment sur la santé, l'éducation, l'environnement ou la sécurité des populations. Mes collègues compléteront ces cours propos liminaire mais à nos yeux le chantier du logement est prioritaire, immense, est absolument vital pour nous outre-mer. Merci cher collègue. La parole est à président Guillaume Gontard, au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer pour cinq minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. Monsieur le président de la délégation. Le président Artano vous a présenté à l'instant succinctement les axes majeurs du riche. Rapport de la délégation outre-mer reconstruire la politique du logement outre-mer. Mais excellent apportèrent Micheline Jacques et Victorien Lurel que je remercie de leur confiance pour m'exprimer au nom de la délégation.-- Mes collègues donc vous préciseront nos travaux et nos propositions sur les 2 premières parties du rapport refonder les cas de la politique du logement outre-mer qu'il s'agisse des financements, mais également du besoin de penser une politique plus adaptées à chaque territoire et plus en appui des collectivités locales et puis faciliter l'accès des populations à un habitat décent en diminuant le coût des opérations immobilières notamment via une adaptation normative mais aussi en résorbant l'habitat indigne, en réhabilitant parc existant et en accélérant la construction de logements sociaux. Pour ma part je me concentrerai sur la liste sur la 3ème partie du rapport que j'ai plus précises, plus directement piloté au delà des difficultés structurelles dont les constats sont posés dans ce rapport l'habitat dans les outre-mer peut être un modèle d'adaptation et d'innovation pour répondre au niveau des filles de la politique du logement. Ceci pour 3 raisons principales, d'abord les Outre-mer sont de véritables laboratoires des évolutions des besoins de logements et des modes d'habitats, ensuite ils sont déjà un terrain d'expérimentation pour l'adaptation de dispositifs et de procédures innovant. Enfin les outre-mer ont un formidable potentiel de systèmes constructifs locaux adaptés aux nouveaux défis du logement comme le réchauffement climatique qu'il conviendrait surtout de mieux promouvoir et mutualisée. Dit autrement, comment sortir de la standardisation de la production de logements et du tout béton. Comment réduire les coûts de construction, tout en améliorant la qualité. Comment limiter la dépendance énergétique des logements et respecter les ambitions de la stratégie bas-carbone. Comment renforcer la religion du bâti face aux catastrophes naturelles. Comment encore construire pour s'adapter aux évolutions démographiques, notamment le vieillissement. Notamment exemple le vieillissement et au mode de vie, tournée vers le plein air tout cela en favorisant les économies locales. La bonne nouvelle c'est que la réponse à tous ces défis et presque unique. Développé une filière locale du bâtiment. S'appuyant sur le savoir-faire des architectes ultramarins notamment la mémoire de l'habitat vernaculaire sur des matériaux locaux et bio-sourcés le bois le bambou la brique la terre. Et j'en passe pour bâtir des nouvelles formes d'habitat léger ouvert moins gourmands en énergie et plus résilients face aux risques climatiques. À rebours de notre jacobinisme historique. L'enjeu est de s'adapter aux spécificités de chaque territoire ultramarin. Cela passe naturellement par un assouplissement ou une adaptation des normes en vigueur que le rapport détaille. Pour ne prendre qu'un exemple, il est indispensable de faciliter la certification des matériaux biosourcés venant des pays voisins, de nos Drôme. Pour leur permettre de raccourcir les circuits d'approvisionnement cela passe également par une meilleure utilisation des financements publics pour financer notamment les éco-quartiers. Cela doit permettre de penser un habitat et je pense notamment à l'habitat social plus ouvert et inclusif avec des espaces extérieurs et des espaces verts, favorisant une meilleure aération une diminution des frais de climatisation et permettant un mode de vie souvent plus collectif qu'en métropole et tourné vers l'extérieur. S'agissant des risques sismiques et cycloniques. La problématique est grande l'habitat léger et plus résiliant face au risques sismiques, l'habitant en béton plus résiliant face au risque cyclonique pour concilier les deux deux rester cohérent avec sa philosophie générale. Le rapport suggère de favoriser l'habitat léger et de prévenir le risque cyclonique avec des pièces sécurisées dans des logements ainsi que des refuges collectifs. C'est donc une filière économique complète et complètement Local architecture matériaux majoritairement biosourcés, bureau d'étude Maîtrise d'oeuvre qu'il nous faut développer une filière à la fois pourvoyeuse d'activité économique et d'emploi une filière écologiquement beaucoup plus vertueuses une filière enfin permettant de bâtir mieux Pour ce faire, nous préconisons préconisant l'organisation d'assises pour la construction ultra du tram Marine qui réunirait l'ensemble des acteurs publics et privés et aurait notamment pour objet à la fois de valoriser des initiatives techniques matériaux et expériences locales mutualiser les bonnes pratiques les réussites et le retour d'expérience et enfin proposer une révision des normes de construction et bien sûr bien d'autres choses. Faisons de nos territoires ultramarins. Un laboratoire de l'innovation, écologique et sociale, en matière de logement. Monsieur le Ministre, nous, nous n'attendons que votre signal. Merci. Merci cher collègue. Dans la discussion générale donc. La parole est à Madame Marie-Claude variations pour le groupe CRCE pour cinq minutes. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre. Monsieur le président de la délégation, chers collègues. Nous voici réunis pour discuter d'un sujet important et dont les réponses ne sont toujours pas la hauteur des besoins. Le logement c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous les demandes explosent après précarité la précarité grandissante, la population a besoin de compter sur une réelle politique du logement pour faire face à l'ensemble des enjeux. C'est d'autant plus vrai en mer ou trop souvent les problématiques métropolitaines s'il trouve exacerbée. L'échec du premier plan logement outre-mer entre 2015 et 2019 témoigne d'une fait une inefficacité du gouvernement de porter collectivement avec tous les acteurs des territoires des réponses locales et concrètes face à la diversité spécificités de chaque territoire ultramarin apporter une réponse verticale n'a pas été la solution. Le second plan logement outre-mer qui a été allongée d'un an afin de prendre en compte la crise sanitaire a comme volonté de faire avec tous les acteurs concernés par la politique du logement en outre-mer les collectivités, les services et déconcentrés les bailleurs, les représentants de locataires et tant d'autres. Est-ce la réalité dans les faits, la route est encore longue et les difficultés sont encore présentes, 80% de la population. Un maire est éligible au logement social alors qu'ils constituent uniquement 18% du parc immobilier. Ce taux d'éligibilité est supérieur à la moyenne nationale, qui tourne autour de 73%. Le 27e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal logement revenez sur la situation en Outre-mer l'État n'est toujours pas au rendez-vous. Plus un seul sans disait le président de la République en 2017, aujourd'hui. Le nombre de sans-domicile-fixe explose l'accès au logement n'est pas garanti pour toutes et tous la pauvreté en Outre-mer et 2 à 5 fois plus élevé qu'en France métropolitaine, le droit de vivre dignement et condamné et cela est d'autant plus frappant à Mayotte et en Guyane, les loyers sont chers. L'accès au logement devient difficile face à des revenus là encore inférieur à la moyenne nationale. Il faut accompagner nos concitoyens et on ne peut imaginer une politique du logement sans prendre en compte la détresse sociale. Alors Monsieur le ministre, il faut élaborer une réelle stratégie autour du logement une stratégie efficace efficiente pour répondre à ces problématiques y compris en outre-mer les associations nous interpelle il faut des produire 15.000 logements par an pour répondre à la demande globale des territoires ultramarins. Aujourd'hui nous n'arrivons guerre atteindre les 10.000 par an, fixé par la loi de programmation relative à l'égalité réelle à l'outre-mer l'habitat indigne représente 13% du parc. Immobilier en outre-mer rien qu'à Mayotte, il y a autant de personnes vivant dans un bidonville que dans tout l'hexagone. L'habitat privé est également fortement dégradé et des moyens sont indispensables pour accompagner les réhabilitations et les opérations de désamiantage. La rareté du foncier. Le réchauffement climatique, la croissance démographique sont des enjeux centraux à intégrer pour permettre à chaque habitant d'outre-mer de vivre dignement. La réponse à ces objectifs doit passer par des discussions et des échanges en associant tous les acteurs liés à la politique du logement en outre-mer des territoires ultramarins font partie intégrante de la République et doivent être représentés dans chaque instance nationale et donc pour les questions de logement également les dispositifs existants doivent être plus lisible, plus transparent, afin que chacune et chacun. Puissent accéder à ses droits concernant le logement, la propriété les travaux. Le développement de l'ingénierie l'eau. Karl mais aussi de l'accompagnement de l'État sont importants, il faut accompagner les collectivités territoriales en leur octroyant plus de moyens humains et financiers pour qu'elle puisse assurer leur mission de service public, l'accompagnement des bailleurs sociaux bien évidemment est également important pour protéger le parc social et les locataires et développer l'offre. J'espère fortement que ce débat et le travail engagé sur le sujet permettront d'avancer sur la politique du logement en France métropolitaine aussi et et en outre-mer le Conseil interministériel des outre-mer qui se tiendra au printemps sera un moment décisif pour les territoires ultramarins. Nous espérons que les annonces seront à la hauteur des engagements pris par votre gouvernement. Monsieur le Ministre, mais surtout à la hauteur des besoins. Car la détresse est grande. Monsieur le Ministre, je termine. En vous posant cette question parviendrez-vous à atteindre l'objectif des 15.000 logements par an en outre-mer malgré la baisse drastique des moyens alloués. Merci. Madame la sénatrice. Autant je partage. Votre analyse sur les 10 sur les besoins. Et on y reviendra tout au long de la soirée sur ce qui ne va pas autant je n'approuve pas l'idée que le seul responsable c'est le gouvernement. Nous sommes tous collectivement responsables. Nous sommes tous collectivement responsables. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de territoires sur lesquels le gouvernement n'a aucune compétence en matière de logement, n'est-ce pas Monsieur Artano mais on va y revenir hein. Mais on va y revenir. Mais je réponds à votre question. Oui, nous devons changer.-- Et j'ai décidé de proposer à tous non pas un plan 3 mais un objectif logement pour la période qui vient. Ce coup-ci signé par les collectivités locales. Signé par les présidents d'association des maires territorialisée. Dans chaque. Chacun des territoires des îles ou territoires. Aussi, pas les représentants des organismes HLM. Il nous faut changer de méthode. C'est ça l'objectif. Et cela devrait sortir non pas sur un plan de trois mais sur un objectif logement partager avec tous les partenaires, ça c'est clair. J'ai un problème et celui, je vous dirai celui-là. J'ai un problème foncier.-- Et un problème de simplification, effectivement dans le cadre du Chiome suite. Suite à l'appel de Fort-de-France et suite à la soirée du 7 septembre. Il y a un certain nombre de données qui me sont revenus, on est en train de les mettre en oeuvre les mettre en route, il faut bien calibrer tout ça parce qu'on ne fera pas 500 mesure il faut faire celle qui. Impacte le plus notre capacité à faire ensemble du logement. après on y reviendra sûrement dans la soirée. J'ai un problème de foncier. Foncier pour lesquels je le dis très simplement, les collectivités locales largement propriétaires de foncier disponible seront sollicités fermement.

La seule chose qui a changé, sous l'impulsion du président de la République aussi le maintenant de le faire ensemble.-- Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous venez de le dire le plan hein n'a pas tenu son objectif de construire et de réhabiliter 10.000 logements par an malgré les outils mobilisés les plans successifs, le constat est sans équivoque, le secteur du logement reste en crise sur l'ensemble des territoires ultramarins. Nous n'avons pas encore le bilan détaillé du plan de et nous souhaitons vivement pouvoir en lire les réalisations, les perspectives, vous venez de les donner. Monsieur le Ministre. En clair, avons-nous vraiment reculer sur le nombre d'habitat indigne encore trop important dans les Drom alors même que la salle l'insalubrité impacte la santé physique et mentale des publics vulnérables. Je pense aux habitants infesté de moustiques à les de la d'un à l'épidémie de la dame qui en a suivi par exemple à la Réunion et qui sévit encore à la déscolarisation précoce la procureure précarisation des femmes battues qu'ne retrouve pas un logement social de manière aussi évidente. Alors même qu'on leur on le, on De la même façon. Quels sont les résultats en matière de l'amélioration de l'habitat prisée entre les aides du 1% logement et il y a des moyens financiers, la prime rénovent de l'État et les aides régionales existant, ça existe dans beaucoup de collectivités. Force est de constater que l'éparpillement des dispositifs freine leur mobilisation respective, alors que nous savons qu'il existe des dispositifs. Il y a aussi un autre point de vie vigilance le vieillissement de la population ultramarine particulièrement accéléré aux Antilles qui nécessite un véritable plan stratégique, comme le préconise le rapport Broussy de mai 2021. En 2050, la Martinique sera le département le plus vieux de France, face à ce scénario catastrophe. Ce plan doit être élargie aux autres territoires également touchés par la transition démographique. Nous avons la grosse difficulté avec l'île de la Réunion et Mayotte à côté puisque la Réunion atteindra les un million d'habitants avant même qu'on arrive. L'année 2030 en ce qui concerne le logement de la jeunesse. Tous les acteurs bailleurs sociaux compris reconnaissent qu'elle a de plus en plus de mal à accéder à un logement qu'ils soient jeunes travailleurs ou étudiants le Domiens à des difficultés pour se loger. Je vous donne un chiffre, pour la réunion il y a 1380. Une place pour le Crous alors que nous avons 21.000 étudiants et ce constat n'est pas différent dans les autres départements des territoires ultramarins. Dans les autres outre-mer et vous avez raison, Monsieur le Ministre, ça n'est pas seulement de la faute il y a une incurie collective. Entre. La réserve foncière qui n'a pas été mise en place mais nous savons, nous le constatons, les défis sont nombreux, variés au sifflet dont nous pour une plus grande territorialisation de la politique du logement, vous venez d'en d'en parler car il convient de mieux prendre en compte les particularités de chaque territoire pour mieux répondre aux attentes de la population et des cons cette territorialisation doit aussi passer par une meilleure représentation des outre-mer dans les instances nationales du logement par exemple, le ministère des Outre-mer. Ne siège pas n'est ni membre du conseil d'administration de l'Lana qui n'est pas suffisamment mobilisés dans nos territoires, ni dans celui de la rue et on peut s'interroger sur cette absence, mes chers collègues. Car si nous voulons résorber les habitats indignes si nous reconnaissons l'inadaptation normative rappelé par les collègues dans le secteur du bâtiment, décrié depuis de nombreuses années comme étant l'un des facteurs du renchérissement des coûts de la construction. Si nous reconnaissons exact et effectivement l'exiguïté de la réserve foncière et le manque de financement au niveau du froid qu'il s'agit du froid. Son principal ou du fera-ce donc secondaire. Nous savons qu'aucune collectivité ne pourra avoir de la réserve foncière souvent sur des territoires où il y a des pentes aménager en a ensuite ces ces ces terrains que peuvent mettre à disposition les communes quand il s'agit par exemple pour la réunion des communes D. O. reconnaissons alors qu'un vrai plan Marshall du logement en outre-mer est nécessaire, bien plus qu'un plan 3 et au-delà même de l'augmentation de la LBU car il ne s'agit pas seulement de la ligne budgétaire unique, nous pourrions être de véritables laboratoires à ciel ouvert. Car les outre-Outre-mer sont des Terres d'innovation et d'expérimentation, le répète souvent les grandes tendances de l'habitat de demain. Ils sont déjà perceptibles et identifié avec l'utilisation du bambou. Ou du chance par exemple avec les galettes de de chambres qui peuvent servir à la construction comme l'utilisation du bois de de Gaulle y aviez ou du crypto-Maria à la Réunion. Mais aussi dans d'autres territoires. J'ai pu le voir et je je je fais je peux faire aussi allusion au Banga qu'on construit par exemple à Mayotte, et qui peuvent être améliorées fortement pour de l'habitat local nous pourrions développer une filière de recherche et de développement de l'habitat innovant avec de nouveaux matériaux, ce qui constituerait un levier important permettant de mobiliser davantage des financements européens dédié à l'innovation car il y a des lignes budgétaires européens qui sont largement sous-utilisés dans ce domaine de l'habitat à cet égard, le chantier de la performance énergétique des bâtiments constituerait aussi un test. Monsieur le Ministre, ancien en tant qu'ancien président de la creux, vous le savez parce que dans le même ordre d'idée, on pourrait envisager de modifier la RTT ah d'hommes avec tout ce qui touche à la réglementation thermique acoustique et aération avec une obligation d'installer des panneaux en complément des chauffe-eau solaires largement déjà mobilisés à la Réunion par exemple développé le photovoltaïque pourtant à terme à l'autonomie énergétique dans l'ensemble des territoires me semble être de bon aloi aujourd'hui pour améliorer également les habitats indignes que qui sont largement. Présents dans l'ensemble des territoires. Le Sénat a d'ailleurs adopté un amendement qui vise à rendre est de nouveau éligible. Les installations de production d'électricité vous le savez utilisant donc l'énergie radiatif du soleil.-- Quant au plan de réhabilitation des logements sociaux ancien il y a bien un plan avec des moyens de l'État qui ont été alloués. Les bailleurs en compte malgré tout de grosses difficultés financières pour répondre à leurs obligations. Vous l'aurez donc compris et on l'a dit avant moi. Au cours de ces dernières décennies. Nous ne sommes pas parvenus à traiter le mal logement dans les outre-mer ni à corriger l'accroissement des disparités car les prix immobiliers ont doublé de manière disproportionnée par rapport à ceux des niveaux de revenus et il est de plus en plus difficile de devenir propriétaire. Quand vous habitez sur un des territoires ultramarins, en clair tout cela dessine les contours de territoire inégalitaire. C'est pour ça que le logement, le mal-logement. La politique du logement social reste un gros problème et un défi à relever pour la population et pour l'ensemble de nos territoires et également pour les mères qui ont à faire face à à ce problème du logement et ces territoires inégalitaire sur le critère de la capacité à constituer un Patrimoine. Pour les Domiens. Et à accéder un cadre de vie adaptés aux aspirations à la diversité des compositions familiales et vécu de manière très forte par des populations qui se sentent oubliés ces disparités fortes sur les marchés. Vous en avez parlé aux conséquences directes sur la capacité d'accès au logement des ménages pose également la question du creusement et c'est pour ça que les territoires ultramarins se sentent parfois les grands oubliés de la politique nationale, alors même que nous savons que des moyens financiers sont mises en place et donc vous aurez compris que les les débats reste ouvert. Et je ne parle pas de la loi SRU ou de l'application de la loi than. Comment appliquera-t-on la loi dans dans les Dom. Monsieur le Ministre, chers collègues, je plaide, comme vous pour une plus grande. Hector réalisation de la politique du logement et un plan d'urgence que je ne dors plan car un coup afin qu'aucun Domiens ne soit laissé sur le bord du chemin.

Elle est recevoir la la la directrice générale de l'ANRU dans les semaines qui viennent. Par exemple sur le sujet, pourquoi ne construit ne sont pas de logement HLM en Z PNRU ça veut dire qu'on en construit plus à l'outre- mer en réunion. On va changer ça. Donc je veux dire, essayons les. D'abord il y a les problèmes généraux et puis après on les territorialisée. C'est tout ce que je veux faire dans ce. La suite du Plot mais que je vais l'appeler objectif logement pour l'outre-mer objectif logement ensemble.

C'est comme ça qu'on me l'a décrit, mais vous allez m'en, m'en parler en tout cas ça prend sur la LBU. J'donc le sujet de qu'est-ce qu'on finance avec la LBU. Il faut qu'on se mette d'accord ensemble et peut-être ne devrait-on pas financer les mêmes choses selon les territoires sur la. Le but, c'est ça la territorialisation quel je je fais attention.-- Il nous faut et c'est un des sujets quand même avoir des organismes HLM plus dynamique.-- Je les aime beaucoup mais ça repose quand même sur. Il nous faut travailler sur la qui ne fait pas tout à fait le job outre-mer hein. Le nombre de logements vacants à réhabiliter est considérable. Alors j'ai invité le président de l'à venir me voir avec la directrice. Pour qu'qui rentrent dans le système pour l'instant ils sont un peu. Ailleurs, on va dire hein non, essayons de bien cerner les questions de bien cerner les priorités. De tirer territorialiser les priorités parce qu'elles sont pas les mêmes selon les territoires. C'est pas les mêmes hein

Juste sur le fera fut Monsieur le Ministre, le fera fut est un fonds qui concerne l'aménagement et c'est souvent ce qui coûte le plus cher. Alors vous avez raison. On utilise souvent de la la quand on a besoin d'aménager les routes pour faire les logements sociaux mais on pourrait mobiliser fortement le fera fut. Oh oh via les dispositifs européens.-- Si monsieur Stéphane Artano pour le groupe RDSE pour cinq minutes. Monsieur le. Le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il est vrai que ces dernières années. La question du logement a fait de nombreux. Que de nombreux rapports ou d'amendements visant à améliorer le traitement de l'habitat indigne et faciliter la production de logements sociaux, ça a été dit par monsieur le Ministre, mais la situation reste toujours autant préoccupante et contraignante. En effet, force est de constater que leur déclinaison opérationnelle tarde à se concrétiser et les effets à se faire sentir en parlant de réalités territoriales, Monsieur le Ministre, je vais me permettre d'apporter quelques précisions sur les dispositifs relatifs au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon. On application de la loi organique et vous saurez me le rappeler évidemment la compétence en matière de logement appartient à la collectivité, par voie de conséquence par exemple la loi de 1989 sur logement qui est dort public dont les ne l'est pas, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, à travers son schéma territorial d'aménagement d'urbanisme de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon porte un véritable projet d'accompagnement à la rénovation thermique et parallèlement mène un processus d'élaboration d'un programme territoriale de l'habitat. Il est vrai que dans le contexte immobilier tandis que nous connaissons la collectivité souhaite répondre aux besoins de la population. Quant à la pénurie du parc de logements. Les bâtisses sont parfois dégradées tandis que les loyers proposés ainsi que les coûts à l'achat ont fortement augmenté ces dernières années et ne sont plus du tout maîtrisé. Dans ce cadre il est nécessaire de réfléchir à la mise en place d'outils fiscaux sur lesquelles travaille la collectivité contre la vacance et la rétention foncière ainsi que le déploiement d'un système d'aide incitatif à la rénovation argentique avec un focus social et urbanistique. Nous devons aussi étudier la faisabilité de l'instauration d'un code de la construction et de l'habitation. En prenant en compte la reconnaissance des normes pour les matériaux nord-américains. Localement et la pratique dominante de l'auto-construction. Afin de répondre à ces quelques problématiques. Je souhaite vous interpeller sur 5 thèmes, il pourrait y en avoir d'autres mais au moins 5 thèmes, ce soir, Monsieur le Ministre. Tout d'abord concernant la réactivation de la ligne budgétaire unique pour Saint-Pierre-et-Miquelon que vous avez évoquées, je rappelle que ce dispositif a constitué un réel effet de levier pour la création d'une offre de marché locatif aidé entre 81 et 2015. La réactivation de ce dispositif permettrait d'augmenter rapidement l'offre locative et redonnerait de l'activité par ailleurs au secteur du bâtiment et aux PME de la construction à un coût réduit pour la puissance publique et in fine et pour le particulier. Ensuite, concernant le rôle de l'État dans la politique de logement social sur le territoire. Celui-ci doit être clarifiée, me semble-t-il en matière de financement des résidences sociales et aide personnalisée au logement. Par ailleurs, la collectivité territoriale souhaite que l'État puisse accompagner dans leurs projets de rénovation d'adaptation des personnes en perte d'autonomie ou de handicap. À Saint-Pierre-et-Miquelon et Miquelon à ce jour. Nous n'entrons pas encore dans le Champ d'intervention que vous avez évoqué, monsieur le Ministre de l'Lana. Qui reste malgré tout un partenaire privilégié des collectivités territoriales, dont le développement de leur politique de logement, il nous paraît indiscutable que l'appui méthodologique et les moyens financiers proposés par l'Anaes permettrait à l'archipel de se doter d'une véritable politique de l'habitat. J'en termine au niveau presque de mes questionnements. Regard des objectifs fixés par le gouvernement et je sais que le député Stéphane Lenormand a interrogé le gouvernement récemment à l'Assemblée en matière de consommation d'énergie de rénovation thermique. L'État pourrait-il s'engager à étudier les possibilités d'accompagnement des usagers dans leur projet de rénovation et l'adaptation du logement en tenant compte à la fois sur le plan des financements que d'expertise on appuie au point info énergie, qui a été mis en place sur le territoire et puis 5ème et non des moindres, et vous l'avez évoqué, monsieur le Ministre. Le déplacement du village de Miquelon avec. Les changements climatiques et la montée des eaux, la nécessaire la nécessité de de s'adapter de re-urbanisée de nouvelles zones pour avoir un village à une centaine d'années maintenant, puisque c'est un peu l'objectif que tous les élus se sont fixés avec une initiative lancée par la mienne Miquelon soutenu par l'État, donc le gouvernement et la collectivité territoriale. Effectivement, la question se pose aujourd'hui des moyens financiers qui pourront être mis sur la table pour pouvoir accompagner la mise en oeuvre des réseaux de la nouvelle zone à urbaniser. Et si vous pouvez nous apporter une reconfirmé, Monsieur le Ministre, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, je pense que tous les habitants de l'archipel, notamment ceux de Miquelon et les jeunes qui voudraient y revenir s'installer. Serait heureux d'entendre cet engagement de l'État. Évidemment que je saurai apprécie à sa juste valeur de manière globale sur la compétence logement et je le dis en anticipant un petit peu il serait je pense inacceptable de s'entendre dire je dis tel que je le pense que cette compétence logement de la collectivité, l'oblige à elle seule à faire face à à celle-ci à se débrouiller seuls. Ce que nous demandons. Monsieur le Ministre. Ce sont des moyens financiers on investissements. On soutien du conseil territorial, ce que nous avons dit d'ailleurs à la Première ministre tout récemment pour qu'on puisse donner une impulsion en terme de d'effet de levier de construction locative sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous savez, on ne parle pas des mêmes effets de levier que sur d'autres territoires ultramarins et les moyens financiers à mobiliser sont pas si énormes que ça si on s'y met tous un peu et ce qu'on demande en réalité c'est un véritable partenariat, d'ailleurs c'est un peu ce que l'État vient de faire en Guadeloupe, avec un soutien massif. Nous l'avons vu au dernier budget et ça a été saluée de 20 millions d'euros pour redresser notamment les finances du syndicat mixte d'eau et assainissement alors qu'on ne peut pas dire que l'État et des compétences en matière d'eau et assainissement. Mais je salue l'initiative et l'investissement de l'État et je suis persuadé qu'il s'agit là d'un c'est de d'Intelligence collective et je suis persuadé également que nous saurons trouver cette voix à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Monsieur le sénateur Artano. Vous savez combien Saint Pierre est chère à mon coeur. Et j'y retournerai, je pense en mars avril quelques quelques réponses simples.-- Oui la compétence logement est à la collectivité et à ce titre l'ANRU là a la LBU et les aides à la Pierre ne s'applique pas. Faut changer ça. Dans une large le monde tel qu'il est à 6000 habitants. On n'arrive pas à voir tout seul avec leur financement. On ne peut pas avoir les mêmes services.

De l'appel de Fort-de-France de modifier soit dans le siom manière institutionnelle pour qu'on puisse intervenir sans. Et ça qui est important. Sans vouloir prendre la compétence qui est la vôtre, mais simplement de nous donner les moyens de vous aider, c'est ça qui est en cause d'ailleurs depuis 2017 à titre dérogatoire. Vous l'avez dit-elle bu finance en partie le logement à Saint-Pierre-et-Miquelon. On va continuer à Didier rogatoire il y a pas de raison de s'arrêter. Mais il nous faut aller vers cette. Responsabilisation différenciation et le débat entamé. Va aboutir. J'entends présenté monsieur le ministre de l'Intérieur, des Outre-mer. En juillet, pour le présenter ensemble en septembre à madame, la Première ministre et au président de la République tout ce volet institutionnel appréciable hein qui qui méritent des changements institutionnels.-- Un mot sur le. Un pont La République a déménagé. Des dizaines de villages.-- Avec les barrages hein notamment avec les les les barrages hydrauliques. Là c'est plus simple je confirme pour avoir travaillé en prévision de.-- Cette réunion de ce soir avec la DG PR la DGPN financera à 100 pour %. Les dépenses individuelles. La question c'est que est-ce qu'on donne le l'aide directement.-- Aux individus hein c'est le fonds Barnier qui joue à plein et qui a de l'argent ou est-ce qu'on essaye de centraliser.-- Ensemble avec monsieur le mot sein de l'État pour savoir si en plus on finance les investissements collectifs c'est ça c'est le sujet de ma prochaine visite au printemps chez vous, monsieur le député.-- Merci la parole est à Madame Micheline Jacques pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, vous le savez, il n'y a pas de politique publique efficace sans cadre normatif adapté. Cette problématique est au coeur des travaux de la délégation sénatoriale aux outre-mer et c'est une approche qui me tient à coeur. En effet, au cours des auditions en vue du rapport logement trop de trop nombreux freins normatif à la production de logements nous ont été rapportés. Or une bonne adaptation permettrait de répondre certes au défi de la production mais aussi à d'autres enjeux. Ils sont notamment environnementaux et peuvent aussi constituer des leviers de production de valeur à laquelle je vous sais Monsieur le Ministre, particulièrement attaché. Comment comprendre que la Guyane ne puisse apporter de bois de charpente du Brésil, mais qu'elles doivent le faire venir de Scandinavie à l'heure du renchérissement des coûts d'énergie fossile et des objectifs de les carbone ation. Cette situation est l'illustration même de l'inadaptation normative. La Guyane pourra également fournir davantage bois la Guadeloupe et à la Martinique. Sachant en outre qu'elle produit des arbres disposant de solides qualités anti-thermiques.-- Autre exemple à Mayotte. L'entrée en vigueur de nouvelles normes pour les portes de garage. Ah je cite entraîné la destruction de toute une partie de l'artisanat local. Voilà un autre exemple de normes qui se concentrant sur l'objectif de sécurité occultes. Les dommages collatéraux qu'elle génère. Il convient désormais au contraire d'évaluer de manière plus globale, l'impact d'normes pour renforcer ce qui pourrait être fragilisé, là encore la protection des savoir-faire locaux peut constituer une formidable source d'innovation tout en répondant à plusieurs enjeux. De fait, la part de recherche et de développement est encore très faible dans les Outre-mer et offre un potentiel de croissance colossale notamment pour l'adaptation des matériaux locaux ou régionaux aux contraintes de sécurité, cela pourrait représenter des opportunités de développement, de formation et pourquoi pas d'école d'ingénieur dans chacun des bassins océaniques. J'ai eu l'occasion de le suggérer lors du débat budgétaire. Par ailleurs, le coût des matériaux représente un des principaux freins à la construction et c'est pourquoi notre délégation préconise notamment les échanges transfrontaliers et avec les îles voisines de matériaux, mais aussi de technique, l'arsenal normatif doit mieux prendre en compte les pratiques des pays voisins dans les conditions climatiques ou d'Exposition aux risques naturels sont plus proches de celles des outre-, mer. Comme l'a rappelé le président Artano, la Nouvelle Calédonie a montré la voie avec un chantier d'acclimatation des normes qui s'appuie largement sur la coopération technique régional avec l'Australie. Si son statut lui permet d'en prendre l'initiative et de maîtriser le c'est suce d'adaptation dans les autres collectivités, l'État pourrait être coordonnateur de la même démarche pour les outre-mer. Elle plaide aussi le plus plusieurs années pour la tenue d'Assises de la construction outre-mer qui favoriserait par surcroît. L'échange de bonnes pratiques. Compte tenu de son expérience. C'est une proposition que la délégation a également relayé et que la direction générale des Outre-mer et la DHUP pourrait organiser. Depuis le rapport de la délégation, le BTP outre-mer au pied du mur normatif. On peut noter les efforts de la part des organismes et administrations producteur de normes techniques. Toutefois il reste encore beaucoup à faire pour territorialisée la certification, les échanges d'informations entre territoires et surtout la production du cadre normatif afin qu'ils ne soient plus essentiellement pensé depuis la métropole, enfin je ne saurais conclure ce propos sans évoquer l'absence de filières de désamiantage dans les autres maires, ce qui entraîne des coûts considérables des propositions de neutralisation existe. Cela m'amène du reste à évoquer l'intérêt de l'utilisation de matériaux biosourcés au détriment du béton. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, je suis convaincu qu'en ces temps troublés et de contraintes budgétaires. Une approche pragmatique du logement ne peut faire l'économie de sa dimension normative.-- Merci cher collègue. Monsieur le Ministre. Madame la sénatrice, puisque vous représentez Saint-Martin et Saint-Barth. Je voudrais d'abord dire que je compte beaucoup sur les collectivités territoriales pour proposer du logement pour proposer des terrains dont ils sont propriétaires. Pour pouvoir construire des logements pour les fonctionnaires. Moi je m'engage à maintien. Si vous me donnez me proposer le proposer des terrains à bail emphytéotique de 60 ans a trouvé des investisseurs qui viendront faire du logement pour les fonctionnaires ça vous coûtera pas un sou, ça coûtera un sou à personne et dans 60 ans c'est à vous. Je suis en train d'écrire à chacun des présidents de collectivités pour dire si il veut du logement des fonctionnaires c'est cinq donne du terrain et tout son nom à Saint-Martin comme à Saint Barth. Notamment. Sur. L'énorme je veux d'abord une bonne nouvelle, c'est qu'en 2023 la mise en place en accord mis en place en accord avec la Commission européenne des marquages outre-mer en substitution marquage CE pour favoriser l'approvisionnement dans le bassin c'est pour 2023 de même production de tableaux d'équivalence à la norme pour l'île de famille de matériaux de construction importés des pays limitrophes outre-mer mais vous avez raison sur les normes, il faut y aller. J'attends et je me suis fâché contre les artisans du club de parce que je trouve que ça ne va pas assez vite, il y a un certain nombre de normes qui vont sortir en 2023 normalement André avancer. Pour le reste, on va lancer dans le cas du FIOM et enfin je suis en discussion avec mes partenaires, mes amis. Hein, hein d'Espagne et du Portugal au niveau des rues. On va faire une réunion à Madrid j'espère rapidement pour essayer d'aller vers une révision Tea Party 349 du traité pour balayer toutes ces normes qui en matière de logement, mais aussi sur d'autres sujets sont un peu bloquant sur. Procéder sur ce qu'on a fermé, il faut y faire attention. L'Europe nous amène beaucoup et donc. On est sur un chemin de crête. Les RUP ça amène beaucoup d'argent et c'est aussi beaucoup de contraintes. Donc c'est ça le chemin qu'il faut trouver, c'est toute l'objet des discussions institutionnelles. Que je mène et je vais d'ailleurs cette semaine à la fois à Martin. Et en Guyane,

Monsieur le Ministre, je voulais juste vous vous préciser que Jean ne représente que la collectivité de Saint-Barthélemy météo. Par conséquent je transmettrai votre réponse au président à vie Merci la parole est à monsieur Pierre Jean Verzeaux laine pour le groupe les indépendants pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La crise du logement dans les outre-mer constituent un problème grave persistant. La question du logement est au centre des attentes et des préoccupations des populations ultramarines.-- Les chiffres sont là, dans les départements et les régions d'outre-mer on évalue à 11.110 1000 pardon. Le nombre de locaux impropres à la à l'habitation et présentant pour leur occupant des risques sanitaires ou sécuritaires. En outre, 80% des ménages des Drôme sont éligibles au logement social et 70% au logement très social. Or ce sont seulement 15% des ménages qui accèdent aux logements sociaux. Sur l'île de la Réunion. Ce sont 33.000 familles qui sont dans l'attente d'un logement social. Enfin on compte près de 120.000 logements vacants dans les Drom ce phénomène concerne en particulier les Antilles. Les conditions de vie dans certains de ces territoires sont indignes de la République. C'est pourquoi il est urgent de mener une grande politique publique ambitieuse en faveur du logement en outre-mer on a compris que c'était pas que l'État, c'est aussi les collectivités, les bailleurs sociaux et que les problématiques était différent selon les territoires. Après l'échec du plan logement outre-mer hein qui n'a pas tenu son objectif de construire et réhabiliter 10.000 logements par an. Le 2ème plan outre-mer a été lancé pour les années 2019 2022. Abandonnant la stratégie quantitative du premier plan, le second qui a été prolongé d'un an, présente une nouvelle approche tendant à mieux prendre en compte les spécificités des territoires et les enjeux qualitatifs. Aussi, Monsieur le Ministre quel 1er bilan pouvez-vous nous présenter en matière de construction de logements locatifs sociaux et très sociaux et de logements réservés à des publics ciblés. Quels chiffres, pouvez-vous également nous donner sur l'action du gouvernement menée en faveur de la résorption de l'habitat insalubre.-- Qu'en est-il enfin de la réhabilitation du parc locatif social et de l'accession sociale à la propriété destiné aux ménages sous ces plafonds de ressources.-- Face à l'ampleur de la crise du logement ultramarin qui, faute d'une véritable politique volontariste de l'État et depuis longtemps ne pourra que s'aggraver et enfin d'anticiper l'après-plan, la délégation sénatoriale outre-mer a recommandé au gouvernement dans ce rapport d'information datant de juillet 2021 la mise en oeuvre d'une action territorialisée et adaptée aux facteurs économiques, environnementaux et humains des Outre-mer. À cet égard il paraît. Nous en avons parlé pertinent que cette territorialisation se traduisent notamment par une véritable représentation des outre-mer dans chacune des instances nationales du logement. En effet, le ministère des Outre-mer n'est membre ni du conseil d'administration de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, ni de celui de l'Agence nationale de l'habitat. De même, on peut regretter l'absence d'un parlementaire ultramarins au conseil d'administration de l'. Enfin il paraîtrait approprié que les agences nationales telles que l'Action logement ou la banque des territoires désigne des référents locaux au sein de chaque territoire ultramarin. Monsieur le Ministre, mes chers collègues pour être efficiente, la politique du logement dans les outre-mer requiert des objectifs concrets et territorialement adaptée, elle nécessite également une volonté forte de l'État et une ambition du sur mesure. Elle exige aussi un pilotage au plus près des acteurs locaux. Merci de votre attention et vos réponses. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. dans ce que j'ai appelé l'objectif logement ensemble. D'évaluation quantitative. De ce qu'il a à faire, c'est juste un truc pour se retaper derrière hein le ski à faire ensemble, c'est le plus possible, on a de la marge, plus on peut en faire plus, on y arrivera je confirme donc cet objectif qui vous me permettez de clarifier ma pensée, que la suite du club de c'est un document dit objectif logement outre- mer signé par l'ensemble des partis et pas simplement par l'appareil d'État. C'est clair et notamment. J'ai un sujet grave qui est lino que vous avez soulevées c'est l'inoccupation d'un certain nombre de logements qui sont vacants et qui permettrait de loger des dizaines de milliers de personnes. Donc il nous faut dans le cadre du travail avec Je l'ai dit tout à l'heure je vais rencontrer le président et le directeur ou la directrice de la dans les jours qui viennent. D'avoir quelque chose de fort.-- Quant au rétablissement de l'aide à l'accession sociale a sorti de l'insalubrité. Dans le cas du PLF 2020. On a dit qu'on pouvait lutter contre l'habitat indigne. On a multiplié par 2. La mobilisation de crédit LBU. Destiné aux opérations de résorption de l'habitat indigne, entre 2019 et 2000 n'est à 32 millions. Mais je voudrais globalement tout ce que vous dites, vous avez raison.-- Mais je crois qu'il faut avoir cette vision d'ensemble que chacun appelle hein que chacun à peine.-- Sans se dit on fait. D'un plan logement outre-mer et Tato étatique. Hein mais d'un plan logement outre-d'un n'Objectif logement outre-mer. Qui soit à la fois signé par tout le monde, qui est une vision globale d'une part et qui a pris, territoire par territoire, dit là où il faut porter les efforts, ce n'est pas vrai qu'on fait les mêmes efforts qu'il faille faire les mêmes efforts hein à la Réunion qu'à Mayotte, à Saint-, Pierre qu'en Martinique. C'est ce qu'on va essayer de faire et je pense qu'on va y arriver si tout le monde accepte de signer ce débat, il me faut un moi le marin, je m'arrête.-- Merci, vous aurez d'autres occasions de revenir sur le sujet. Monsieur vers Alors la parole est à monsieur Daniel Salmon pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Les problématiques de la politique du logement outre-mer sont nombreuses. Et le très riche. Rapport de la délégation outre-mer dont nous discutons aujourd'hui en brosse un portrait éloquent. Parmi les nombreux sujets soulevés par le rapport et les 77 recommandations qu'il formule dans le temps qu'il mette un parti, j'ai souhaité concentrer mon propos sur la dernière série de recommandations des recommandations relatives aux nécessaires évolutions de la construction pour s'adapter tout à la fois aux besoins des territoires et aux dérèglements climatiques, avec son corollaire de catastrophes naturelles qui n'épargne pas, loin s'en faut. Nos territoires ultramarins. Inventé l'habitat résiliant de demain. Construit à partir de matériaux biosourcés est un impératif. Quand le bâtiment représente les 3 cinquièmes des déchets du pays. Des matériaux produits localement à partir de filières durable. Du bois de la terre de la paille chance de bambou un habitat imaginé par des architectes pour répondre aux besoins spécifiques des territoires. En tenant compte de leur géographie de leur climat des modes de vie de leurs habitants un habitat plus économes en énergie plus résilients face aux catastrophes naturelles qui vont se multiplier. Au-delà des Outre-mer inventé cet habitat de demain est un défi pour l'ensemble du pays. Fidèles à leur tradition décentralisatrice, les écologistes ont toujours plaidé pour la différenciation des territoires, l'adaptation des normes, le renforcement des tissus économiques locaux.-- Ce qui est vrai pour résorber la fracture territoriale en métropole prend une dimension bien supérieur. Dès qu'il s'agit des territoires ultramarins.-- De nombreuses préconisations du rapport ont un intérêt majeur. Elle permettrait de renforcer, de créer des tissus économiques locaux de créer des emplois pour tout le niveau de qualification, de créer de la richesse et de limiter l'exode de la jeunesse ultramarine exode responsable également du vieillissement évoqués dans le rapport.-- Au-delà des nombreux bénéfices écologiques de ses propositions sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Leur mise en oeuvre permettrait de doter les territoires ultramarins d'outils concrets pour prendre à bras le corps le défi du logement dont nous débattons ce soir. Chaque territoire ultramarin dispose de savoir-faire traditionnels qu'il faudrait non seulement sauvegarder mais aussi valorisé.-- Ainsi la renaissance de la filière de la brique de terre comprimée à Mayotte doit ainsi être soutenu et étendu à d'autres expérimentations. Dans tous les territoires les potentialités sont multiples. J'en citerai quelques-unes. Je vous les cite pour vous faire un peu voyagé pas hein des Caraïbes bambou Bagasse vétiver Fall cata Amaranth appelé aussi bouillant bois violet Angélique Gaillac Wakapou pas L'exemple de l'Écomusée est effaré Natura amoraux et Moorea en Polynésie, Polynésie française conçue pour mettre en avant le bois et le style locale doit être érigée en modèle avec les matériaux biosourcés c'est l'habitat vernaculaire qu'il faut réhabiliter. Partout, une solution alternative existe, il faut substituer au béton, des matériaux locaux moins onéreux, plus vertueux et beaucoup plus efficace. Compte tenu des conditions climatiques et résiste mieux souvent à l'humidité, la salinité de l'air plus efficace également pour concevoir des logements plus aéré et diminuant les besoins en climatisation mieux isoler pour limiter les besoins thermiques plus efficace également. Face au risque sismique. Si le béton a d'indéniables qualités et il ne faut pas le nier s'il résiste notamment mieux au risque cyclonique c'est également une ressource non renouvelable et. Des alternatives doivent être trouvées pour limiter son usage au strict nécessaire comme les auteurs du rapport. Nous pensons qu'il faut plutôt privilégier les techniques locales et déjà expérimenté, plutôt que de durcir la réglementation para-cyclonique. Les architectes auditionnées ont rappelé qu'il savait concilier les différents risques dans la conception de l'habitation mais aussi proposer des solutions de refuge adaptés. Plus largement, nous sommes entièrement favorable à la promotion d'une architecture bioclimatique performante reposant sur des savoir-faire traditionnels sublimée par les connaissances de notre siècle. À ce titre, comme le suggère le rapport les territoires ultramarins sont et peuvent être davantage encore de véritables laboratoires à ciel ouvert des Terres d'innovation et d'expérimentation.-- Considérant les besoins de logements neufs revint 20 trouvera en outre-mer une application plus massive proportionnellement qu'en métropole. faisons de nos territoires ultramarins. Le modèle de nos nouvelles ambitions écologiques en matière de construction en associant matériaux naturels et production d'énergie renouvelable. On pourra ainsi constater que construction vertueuse confort de vie et développement économique se conjugue pour le mieux. ira tout ira ainsi de mieux en mieux, je vous remercie. ne saurait être maire architectes et constructeurs. Je suis d'accord avec vous à 100 pour % à une réserve près, je sais pas si avec ses méthodes on arrivera à faire 80.000 logements sociaux d'urgence et on parce déjà 5000 ce serait pas mal. 80.000 logements sociaux d'urgence qui est le besoin actuel. Mais ce que vous dites monsieur le sénateur. C'est aux maires qu'il faut le dire, c'est aux architectes qu'il faut le dire. Ce n'est pas le ministère de lui en charge de l'outre-mer qui délivrent les permis de construire. Ce n'est pas le ministère de l'outre-mer qui définit les plats de ces. Bâtiments que vous appelez de vos voeux et que j'appelle aussi de mes voeux. Donc on va essayer de faire de la pub. Mais au-delà de la pub. Qu'est ce que vous voulez qu'on fasse de plus. Hein. Alors on va planifier tout ça comme sur le bioéthanol dont je parlais l'autre jour spatiale assemblée ou ici au Sénat, il faut qu'on progresse tous ensemble et je pense que dans cet objectif. Logement, il faudra mettre un paragraphe assez fort hein assez fort pour inciter tout le monde à aller dans ce sens mais en la matière. Je pas passé malheureusement ou heureusement tout compte procéder que par des incitations vis-à-vis des élus locaux.-- Merci monsieur le ministre, Monsieur Salmon. Oui, merci Monsieur le Président, juste pour répondre, Monsieur le Ministre, je pense que ah peut quand même faire un certain nombre de choses, ne serait-ce que pour organiser les filières pour faire de la formation et aussi travailler très clairement sur le côté normatif. Il y a des normes qui sont vous le savez bien très bloquant de vous l'évoquiez tout à l'heure et il faut à enfin arriver à faire des évolutions de l'assouplissement pour qu'il y ait des expérimentations dans ces territoires d'outre-mer merci.-- Merci, cher collègue, la parole est à Marie-. Laure Phinéra Horse, pour le groupe RDPI pour six minutes.--

Monsieur le président. Bonsoir Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La délégation sénatoriale aux outre-mer a publié il y a tout juste 18 mois, un rapport très intéressant sur la politique du logement dans les outre-mer bien entendu la problématique de l'habitat informel a retenu l'attention de mes collègues et méritait d'être débattue ici dans l'hémicycle aussi je profite de l'occasion pour remercier le président Artano pour cette initiative ainsi que les rapporteurs Gontard Lurel et Jacques pour le travail réalisé. Pour répondre à la problématique du logement en outre-mer le Parlement adopte notamment en novembre 2018 dans le cadre de la loi Elan des dispositions spécifiques à la Guyane et à Mayotte pour lutter contre l'habitat informel, le législateur donner ainsi aux représentant de l'État de Guyane et de Mayotte, le pouvoir d'ordonner aux occupants des habitats informels d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à la démolition des structures dès lors qu'elle présente des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. La nouveauté réside dans le fait que les préfets pouvait ordonner les démolitions sont passés par une décision judiciaire. Nous pouvons le dire la loi Elan a suscité un formidable espoir au sein de nos populations éprouvées par le développement des habitats sans droit ni titre, la Guyane et Mayotte sont confrontés à l'accroissement de l'habitat spontané qui se développe sous la pression démographique, conséquence d'une très forte immigration en Guyane un logement sur quatre a été construit son droit ni titre à. Saint-Laurent-du-Maroni comme une frontalière avec le Suriname l'habitat informel représente 60% des logements aussi dès que la mairie par exemple, envisage un projet de construction, le terrain est occupé, il en est de même pour une opération d'intérêt national, dont la mission première et d'enrayer la dynamique du logement informel et anticiper la démographie galopante en créant près de 30.000 logements d'ici 2030. Paradoxalement, de nombreuses zones d'habitat spontané sont installés sur le foncier appartenant à l'État le 1er propriétaire foncier de Guyane. L'impuissance de certains acteurs ne rassure guère les petits propriétaires qui ont ce désagréable sentiment d'être privés de leurs droits, mais aussi du fruit de leur dur labeur. L'ancienne maire que je suis a fréquemment été confrontée aux difficultés liées à l'occupation illégale de logements et au développement de zones d'habitat informel. L'ancienne maire que je suis a souvent eu à intervenir face à la colère des habitants des propriétaires désabusés par les occupations illégales de certains bâtiments et de nos espaces publics et en tant que maire je devais m'employer à calmer l'exaspération des citoyens face à l'inaction de l'État en 2018, alors même que les parlementaires ici au Sénat discuté des contours de la loi Elan une foule vindicative avait procédé des logements d'une dizaine de familles de squat à Cayenne et nous avons évité de peu un drame alors moi aussi j'avais placé beaucoup d'espoirs dans cette loi. loi. 4 ans après, quel bilan pouvons-nous tirer de cette loi en s'appuyant sur l'article 197 de la loi Elan, le préfet de Guyane et de Mayotte en certes ordonné la démolition de plusieurs zones d'habitat spontané des opérations ont permis de raser des dizaines de squat où se côtoyaient insalubrité misère et insécurité mais nous devons avoir la franchise, l'honnêteté de dire que ces opérations n'ont malheureusement pas eu les résultats se Face à la pression migratoire qui frappe ces deux territoires et à la multiplication des contentieux qui ralentissent procédures plusieurs limites sont à souligner. À Mayotte comme en Guyane, le législateur a voulu, au travers de cette loi faciliter l'expulsion des occupants de terrain sans droit ni titre mais le passage de la théorie à la pratique est bien plus complexe que prévu. En effet, dans un élan humaniste, le législateur a conditionné les expulsions à des propositions de relogement mais les préfectures ne sont pas en mesure de proposer des solutions de relogement famille par conséquent les opérations d'évacuation aboutit systématiquement à la reconstruction de nouvelles zones les habitants errent de squat à un autre j'insisterai donc sur ce point la Guyane n'est pas en mesure de proposer des solutions de relogement aux habitants délogés en raison d'une offre de logements quantitativement insuffisant, la Guyane n'est déjà pas en mesure de répondre à la demande en matière de logement de nos compatriotes et depuis 20 ans l'habitat informel progresse bien plus vite que le logement légale. Par conséquent, je me réjouis de ce débat, mais également de l'examen demandé par notre groupe RDPI de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Nous devons chercher de nouvelles adaptations afin que l'état de droit puisse exercer pleinement en Guyane comme à Mayotte, mais aussi dans tous les territoires face aux occupations illicites. Il n'est pas acceptable que certains territoires de la République continue à livrer. Seul ce combat contre l'habitat informel pour conclure, je voudrais rappeler ces quelques mots de l'ancien président de la République François Mitterrand en déplacement officiel en Guyane, en septembre 1985, il s'était offusqué qu'on continue à lancer des fusées sur fond de bidonvilles près de 40 ans plus tard, les fusées décollent toujours les zones d'habitat informel elle se multiplient à la vitesse d'un lanceur au décollage. Voilà monsieur le ministre et a changé de qui. Plus de 40 ans. Voilà ce que je voulais exprimer ce soir, merci. Madame la sénatrice. Effectivement. Ce qui a changé, c'est une pression migratoire extraordinaire pression migratoire dans je veux dire un mot qui est une. J'allais dire une constante. De la Guyane avec les Haïtiens les sur une Amiens et les. Brésiliens notamment le. Ça c'est ça allais dire la tradition de la Guyane, il y a des accueils qui se font avec ce sujet du logement vous nous avons ne mélangeons pas les deux, il y a nouvelle immigration des afghans, des Syriens, des marocains et des Kurdes se là. Je ne veux pas je dis je ne veux pas qui stationnent autour de la cathédrale et j'ai donné instruction de démolir les tende systématiquement.

Donc il y a ce problème d'immigration qui est là. Je suis un ancien préfet. Et je dois dire que entre ordre et désordre hein. On ne sait pas ce qu'il faut. Non je n'ai jamais expulsé sauf cas grave des gens qu'on ne sait pas relogé complètement et comme vous êtes sur un territoire contraint hein on y arrive pas donc la vérité elle est.-- Sur la construction de logements sociaux sur la construction de logements sur des OIN qui démarre enfin j'ai rencontré ce matin Madame Charles, la maire de Cayenne pour dire que.--

de grâce, on a des problèmes.-- Et et je sais que quand je m'adresse à vous, je, je, on pense la même chose, on ne trahit pas son âme hein on ne trahit pas son âme sur les sujets d'immigration. On ne trahit pas son âme sur les sujets de logement.--

Madame finira Horse non c'est bon. La parole est à Madame. Victoire Jasmin pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour cinq minutes.-- Merci monsieur le président. Monsieur le Président Artano Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la question du logement dans les outre-mer a déjà fait de nombreux débats et demeure pour autant toujours une préoccupation majeure de nos populations, comme cela a été souligné dans le rapport numéro 728 intitulé la politique du logement dans les outre-mer de nos collègues sénateurs quant à Guillaume Micheline Jacques et Victorin Lurel avec de nombreuses recommandations afin de permettre la mise en oeuvre du plan pluriannuel pour favoriser la construction de logements sociaux et résorber l'habitat insalubre. Le premier plan logement outre-mer plan de 2015 à 2019 a été un échec. Ça a été dit la non prise en compte dans nos spécificités locales n'a pas permis de conduire une politique de logement efficace les mesures déployées sans réelle ingénierie locales ont laissé nos territoires avec les mêmes problématiques habitat indigne s'dans creuses friche il n'adéquation entre l'offre et la demande et je ne reviens même pas sur les problématiques liées à l'indivision successorale. L'objectif d'assurer un habitat pour toutes les populations dans leur diversité n'a pas été atteint. La mise en place, diplôme de 2019 2022 a tenté de rattraper le retard accumulé pour résorber l'habitat indigne et construire efficacement sur l'ensemble de l'archipel de façon efficiente. On sait de notre population, ce sont 80% des ménages qui sont éligibles au logement sociaux il y a clairement une inadéquation entre l'offre de logements et les besoins exprimés. Il nous appartient aujourd'hui collectivement de trouver des solutions innovantes pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Sa réponse devront s'inscrire dans l'esprit de la loi 3DS en apportant des solutions différenciées car si nos territoires sont exposés pour la plupart aux risques naturels majeurs, ils font cependant face à des contraintes différentes lié en grande partie à leur position géographique mais aussi à la densité de la population de leur territoire. Plus de 5 ans après la production du rapport des formations le BTP outre-mer au pied du mur normatif. Faire de NOx a un atout de 2017 conduit par nos collègues de la délégation sénatoriale aux outre-mer Éric d'Olivier Karine Claireaux et vivait tu Lopez nous pouvons constater que certaines des recommandations formulées n'ont pas eu de l'application concrète des territoires ultramarins et malheureusement dernièrement nous avons vu avec les différents aléas d'une part Irma et Maria en 2017 mais aussi. Fiona récemment il nous avons vu les dégâts qui ont été causées, Monsieur le Ministre, vous y étiez, vous avez vu ce qu'il avait. Il apparaît indispensable de mieux prendre en compte nos modes de construction pour faire face aux risques naturels majeurs mais aussi de repenser l'aménagement du territoire. La réalité socio-économique de nos populations doit aussi conduire à une réflexion et guider nos actions. Comment permettre au plus grand nombre de ménages d'accéder à la propriété avec des coûts de construction. Dans un contexte d'inflation. Quelles mesures, pouvons-nous prendre pour diminuer nos impacts énergétiques lors de la construction des habitations mais aussi dans leur usage quotidien. L'intervention de nos politiques publiques doivent avoir une résonance sur la dimension sociale, environnementale et économique de la vision stratégique dans laquelle nous devons mener les débats pour les orientations des politiques de logement dans les outre-mer afin qu'elles se suivent à court, moyen et long terme. Des exemples de longévité de construction sont à distinguer et peuvent avoir bien évidemment, l'application de nouvelles normes pour servir de base pour l'adaptation de nos pratiques. La maison par exemple à Marie-Galante maisons. D'habitations en bois édifiées dans le centre-ville de grands bouts de Marie-Galante en 1900. La maison. Maison Coloniale de 1870 en bois situé dans la commune de moules. Ces 2 maisons que je cite, toutes les deux en bois et primé par le Loto du patrimoine pour faciliter leur rénovation éternel par interpelle pardon par leur longévité et leur, leur résistance aux aléas climatiques s'exprimer des modes de construction traditionnelle et des styles architecturaux de l'époque en les adaptant à nos modes de vie d'aujourd'hui hé bien c'est étonnant je efficient et je crois aussi environnementales. La mutualisation des expertises locales sur les modes de construction adaptées aux territoires ultramarins doit faire l'objet d'un véritable projet qui pourrait se traduire c'est un double enjeu. Enfin, je terminerai mon propos en rappelant qu'habiter un logement dans les Drom expose aux aléas climatiques et qu'il est important aussi d'assurer ses habitations. Il nous appartient, Monsieur le Ministre de veiller aussi à la maîtrise des coûts de l'assurance parce que les risques sont importants, mais les coûts sont aussi irréversible quoi qu'elle reçoit et n'entraîne pas forcément

janvier prochain des architectes de la Guadeloupe de la Martinique. Nous ferons un colloque justement sur construire en outre-mer en bois, donc je crois que nous sommes sur le bon chemin. Donc vous avez préconisé un certain nombre de dispositions, je crois que c'est déjà le cas. Merci. Merci, monsieur le Ministre. Merci madame la la députée, madame la sénatrice. De sujets que vous avez évoqué les divisions successoral. J'ai rencontré hier ou avant-hier. L'assemblée des notaires qui faisait un colloque. Vous y étiez. Qui était là si vous étiez non Les notaires et puis de même j'ai rencontré derrière les assureurs hein pour dire attention, vous devez participer à cette rénovation des solutions à apporter au logement outre-mer. Sinon on n'arrivera pas sans vous notamment. C'est tout le problème des successions compliqué. Certes à la Martinique et en Guadeloupe, mais je vous parle pas de Mayotte et de Saint-Martin notamment hein donc sur lesquels il nous faut progresser sur ces solutions division successoral successoral qui bloque complètement le phénomène de même. C'est tout le problème des constructions mise sur les 50 pas géométriques hein donc c'est des sujets sur lesquels on travaille avec les collectivités territoriales régionales notamment, pour aboutir à des solutions. Juste un mot sur les logements vacants. C'est un vrai sujet. Si en occuper la moitié des logements vacants. On y arriverait hein on y arrive oui c'est ça c'est un truc qui me préoccupe. Comment peut-on avoir une crise du logement en Guadeloupe Air Martinique qui perdent 5000 logements pas 5000 Avec des milliers de logements vacants. Il nous faut trouver la solution, il nous faut trouver la solution, c'est ensemble qu'on la trouvera avec les notaires avec les les les assureurs notamment et puis un petit point sur la, la Martinique et dans le même sujet. La Martinique et la Guadeloupe, faut-il ou non relever le revenu minimum pour permettre un certain nombre de gens plutôt âgés qui ont réussi mais d'occuper des logements HLM vacants hein. Moi j'y suis favorable et dit favorable, il faut mettre tout ça au point. Voilà, c'est sur l'habitat individuel adapté évidemment que vous avez raison hein mais je donnerai ma conclusion d'ensemble tout à l'heure.--

Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je tenais à tout d'abord à débuter mon propos en saluant l'initiative de la délégation sénatoriale aux outre-mer. Qui a initié ce débat sur la thématique de la politique du logement outre-mer c'est un sujet fondamental pour les habitants de nos territoires ça prépare une crise du logement sans équivalent et qui méritent que notre assemblée travaille sur cette question plus longuement qu'à la marge d'un projet national ou hexagonales. Et chiffre que je vais vous donner ont déjà été moultes fois prononcé dans cet hémicycle, Monsieur le Ministre, vous les connaissez. Le logement c'est ce que j'ai dit à cette prime. À cette même place le 1er décembre dernier. Tout d'abord un constat saisissant. 80% des ultramarins sont éligibles à un logement social et seulement. 15 ans dispose. C'est d'autant plus préoccupant que nos populations vieillissent et que leurs revenus sont plus faibles que dans l'Hexagone. Il est donc impératif de répondre à la demande de besoins annuels en logements sociaux, estimé entre 9000 et 10.000.-- Autre chiffre alarmant les logements indignes insalubres représente près de 13% du parc de logement dans les outre-mer contre 1,3% dans l'Hexagone pour le seul département de la Réunion. Ce sont plus de 100.000 Réunionnais mal logés. 17.000 logements privés repéré comme insalubre. 25.000 familles réunionnaises primo-accédants, en attente d'un logement social. Toujours à la Réunion, au 30 juin 2022, près de 38.000 demandes de logement social en instance et ce alors qu'à peine 2000 logements ont été livrés en moyenne par an sur ce terrain 5 dernières années. La production logement outre-mer est en crise profonde les plombs hein et de n'ont pas répondu aux attentes et tout le monde en convient. Il est temps de redresser la barre, afin de proposer aux ultramarins une politique de logement ambitieuse efficace. Une fois ce diagnostic posé. Nous devons ensemble, Monsieur le Ministre, proposer des actions concrètes afin d'améliorer la situation. Ces solutions existent, elles sont multiples mais encore faut-il les appliquer. Pour que les crédits de la LBU soit mieux consommer, nous devons tout d'abord mettre en adéquation les financements proposés avec les besoins réels à la Réunion par exemple non seulement les clients et l'été 2 sont construits en homme insuffisant mais aussi à un coût trop élevé. La question de l'adaptation des normes et des matériaux doivent être aussi poser mais c'est vrai Monsieur le Ministre, vous l'avez déjà évoqué la rareté et la cherté du foncier mais aussi le surcoût du prix des matériaux doit nous oblige à changer de logiciel, il faut impérativement accès des financements sur les logements pour les feignants et aussi à des petites surfaces à destination des jeunes ménages et des personnes seules sans une adaptation de l'offre mais aussi de la gouvernance avec une décentralisation accrue de la gestion de des crédits. La LBU ne sera pas mieux consommer ni plus efficace. L'ANRU je veux par ailleurs un rôle important dans nos territoires mais elle doit impérativement revoir ses maquettes financières validé avant la crise sanitaire et économique les conséquences de la crise Covid associé au contexte insulaire ont fait exploser les surcoûts. C'est la difficulté sur laquelle je vous en ai déjà parlé, Monsieur le Ministre, est confronté par exemple la ville de Saint-Pierre à la Réunion. Elle a contractualisé avec l'ANRU en mars 2020, à la veille de la crise Covid et se voit désormais contraint de solliciter une modification du calendrier, ainsi qu'une subvention supplémentaire. Pour pouvoir finaliser son programme de rivaux novation et je vous rappelle ici que ce sont quand même 500 logements qui sont en jeu. Parmi les combats qui restent à mener à gagner. Il a une autre agence qui devrait pouvoir intervenir pleinement dans les Drom et s'agit Anna. c'est vrai qu'on l'en a déjà parlé, il est impératif de rendre les propriétaires occupants ultramarins éligibles aux aides délivrées par cet organisme. Cette disparité entre l'Hexagone et les Outre-mer ne peut plus perdurer. il y a également le déploiement des résidences autonomie attendue depuis longtemps et désormais possible depuis la loi du 21 février 2022 lits dites de loi 3DS enfin notre levier c'est la c'est accompagnée l'auto-réhabilitation des logements par l'occupant certains CCAS mène avec succès cette politique il faut l'encourager et la démultiplier. Le département de la réunion, s'est engagé dans cette voie en doublant le nombre de dossiers d'amélioration de l'habitant en passant de 2000 à 4000 par an. À ce titre je conclurai mon propos en saluant le travail de concertation réalisée par l'association des maires du département de la réunion qui s'est auto-saisi de cette problématique. Elle a mené un travail de fond en auditionnant tous les intervenants et qui a abouti à des propositions concrètes. Je citerai son président Serge Hoareau en disant que cette feuille de route établie par la mdr marque une étape importante mais ce n'est en rien.

J'ai demandé. Anne-Claire Mialot de donner toutes les conventions ANRU sur tout le territoire outre-mer sur lequel il fait effectivement il faut toutes les voir pour être plus efficace. Le temps a passé, on est capable de toutes les revoir c'est beaucoup de travail sur la neige. J'ai le même regard que vous. Notamment à. La Réunion. J'ai dit Madame Mialot rend la, la fin du mois la à la à la Réunion pour voir ce qui se passe sur les jeunes. Vous êtes PNRU hein pour savoir si on peut y faire quand même du logement, il suffit de le décider. Donc sinon on est coincé. Je voudrais vous dire aussi qu'un de mes soucis. C'est de savoir ce qui se passe avec les prix d'Action Logement. Ils vont diminuer leur volume. Pour passer de 300 à 130. Parallèlement, bien sûr, la Caisse des dépôts. Est disponible mais c'est pas le même taux. Donc comment on fait pour harmoniser tout ça et continue à avoir des prix qui soient non plus à 0 45 parce que le taux d'intérêt au. Mais qui ne soit pas à 3 6 et ça le débat notamment la réunion. On a beaucoup de logements sociaux à construire ma réponse.-- Merci. Merci Monsieur le Ministre. D'accord. Écoutez je suspends la séance pour 2 minutes.

La séance est reprise. La parole est à Madame, Catherine Conconne pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. Stéphane Artano. Monsieur le Ministre, j'ai envie de vous dire. Faisons un peu la révolution dans ce domaine-là.-- Où vont le Champ des possibles.-- La première chose à faire c'est d'arrêter de traiter le logement outre-mer dans dans ce vrac dit outre-mer. Le logement est l'expression de la vie des gens, de leur histoire, de leur Patrimoine culturel, on ne vit pas la à. Miquelon. De la même manière qu'on vit à Tahiti ou à Fort-de-France. Donc déjà traité ça dans ce global est un peu gênant et empêche d'avoir une lecture extrêmement. Clairvoyante des situations qui sont totalement différentes les unes des autres.-- C'est pourquoi je vais vous parler avant tout de la Martinique et tant qu'à faire que de la Martinique, parce que c'est le pays que je connais le mieux, et par respect pour mes collègues, je préfère qu'il parle de ceux qui. De ceux qui connaissent le mieux également.-- La réalité à la Martinique n'est pas du tout celle que j'ai pu entendre ce soir décrite. Pas du tout. En 70 ans, il y a eu des efforts extrêmement importants qui ont été faits sur le logement à la Martinique, on peut souhaiter, plus on peut souhaiter mieux l'idéal n'existant pas.-- Mais je suis désolé, je ne suis pas si vieille. Et j'ai vu le progrès porté depuis 70 ans pour un meilleur un mieux vivre des habitants de la Martinique. On est loin. Des Canal Alaric tels qu'on les a connus. On est loin des RH il avec des centaines de logements qu'il fallait résorber. Je rappelle que le 1er lotissement populaire de la Martinique c'est celui d'état civil et qu'il a été construit dans les années 20.

S'il y a bien un paquet.-- Qui pourrait être transférés aux collectivités de chacun de ces pays, c'est bien celui du logement et dans le cadre de l'appel de Fort-de-France. 100% de la politique du logement devrait être aujourd'hui j'ai des par les collectivités locales. Comment peut-on encore imaginer en 2023 qu'on attende la LBU venant de la rue Oudinot pour décider de telle ou telle politique de logement sur place. Donnez-nous les moyens. On saura faire, ne vous inquiétez pas. N'ayez sur ça. Aucune équipe. La 2ème, chose que je voulais vous dire Monsieur le Ministre. Partenariat que l'État bien sûr.-- Il y a des réalités qui sont toutes autres. Et vous avez ouvert le sujet tout à l'heure.-- 20.000 logements vacants aujourd'hui à la Martinique et nous perdons entre 4 4500 et 5000 habitants. Le pays est passé de 400.000 habitants a aujourd'hui moins de 350.000 habitants que fait tontes, c'est 20.000 logements vides. J'ai décidé, Monsieur le Ministre, si vous voulez on peut reparler des idées qui ne passe pas par la spoliation de la propriété. Bien au contraire mais qui pourrait redonner vie à ces fantômes.-- Que sont devenus aujourd'hui certains quartiers, certaines villes certaines rues certaines communes dont certaines ont plus de 60% de leur logement devenu vacant. Qu'est-ce qu'on en fait. Faut les occuper, il faut les rois mais.-- Parce qu'on va pas continuer sur 1100 km2 à construire des barreaux de HLM éternellement. J'ai presque envie de dire, Stop.-- Stop, on a plus bouffée d'ailleurs on n'a plus la attire bouffer. Donc aujourd'hui on est face à une politique publique concernant la Martinique. Qui doit être menée dans la dentelle. On est plus dans les constructions de grands ensembles con comme on a pu fait aujourd'hui les choses doivent être faites dans la dentelle densifier les les centres bourgs réoccupées ces logements vacants et ça demande qu'on ait un travail ensemble à faire pour pouvoir pallier au mieux à la réalité de chaque de ces pays et arrêter d'être noyé dans un fracas. J'ai entendu des choses ce soit mais je suis désolé c'est pas la Martinique.-- je, je me suis pas senti concerné donc au centre nous chaque sur nos territoires sur nos réalités et travaillons dans la dentelle de manière extrêmement précise. Et pour terminer, Monsieur le Ministre, vous savez que je suis une adepte de la responsabilité. Donc j'insiste encore certainement que dans le cas de l'appel à Fort de France. Il y a certainement des choses extrêmement pragmatique à faire et le logement pour être un ex-une excellente illustration de cette volonté de responsabilité. Je vois mes Madame la sénatrice. Pour répondre à votre appel sur ce qu'est le logement. Je dire ce que je dirais pas aux sénateurs Lurel tout à l'heure d'humanité. Née à partir de la conscience d'un toit. Qui crée le lieu de l'esprit humain sous le ciel et qui marque la première identité et le 1er refuse de chacun de chacun. C'est ce que j'essaie de croire. C'est ce que je crois et je voudrais faire participer toutes mes administration tout l'appareil d'État à cette croyance et à cette fois. 2ème sujet. Non une vision globale, je crois avoir déjà répandu sur on arrête le plan 3 et on fait un objectif logement territorialisée, avec des principes effectivement et je suis très heureux que vous vous sentiez pas concernés par ce qu'on essaye de faire à Mayotte hein qui ce intellectuellement et en tant que représentant de la nation, bien évidemment, mais les choses doivent être séparés doivent être séparés donc la dessus je je je vous suis. Je vous suis aussi sur. Logement vacants mais j'ai pas de solution pour l'instant faut y réfléchir et puis je reviens sur l'appel de Fort de France et ce que j'appelle moi le 7 septembre. Chacun son maître. là aussi dentelle il y a pas de réponse unique.-- Pour tous les territoires.-- J'ajoute sur le redis. Que dans un 1er temps et je recevrai tous les parlementaires des outre-mer et les parlementaires des délégations outre-mer qui ne sont pas tout à fait les mêmes choses vers 24 ou le 25 janvier pour vous exposer pour exposer ce que je crois être la feuille de route qu'on va partager. Sur cet appel de fonds de France ou cette soirée du 7 septembre.-- Tout est ouvert, tout est ouvert. Attention cependant. À ne pas se aller se laisser aller à Givet machin il faut bien cadré tout ça il faut bien cadré tout ça quand on parle par exemple de, d'autonomie, c'est un terme que j'aime pas parce que personne n'est autonome et tout le monde travaille ensemble, mais peu importe hein il y a tout de suite la notion des recettes de la fiscalité de l'octroi de mer tout ça est ensemble. J'ai donc. Eu l'autorisation, même la demande de mes autorités supérieures. Pour essayer d'aboutir.-- Vers la fin du mois de juillet et je rencontrent chacun des présidents de collectivités signataires, c'est pour ça d'ailleurs que je me rends.

Un coconne 30 secondes. Oui, monsieur le Ministre, mais je crois que nous sommes d'accord. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bienvenue, bienvenue puisque vous partez à la Martinique demain donc d'ores et déjà bienvenue au plus beau pays du monde la Martinique. Merci cher collègue. Pour cette publicité. La parole est à madame Annick Petrus pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes.-- Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je souhaiterais avant toute chose remercie la délégation des outre-mer et son président Monsieur Stéphane Artano pour cette initiative qui permettent à nos territoires d'outre-mer de débats Tsuno ressemblances et nos différences. Nous le savons tous les territoires ne sont pas régis par les mêmes statuts et selon que nous soyons régi par l'article 73 ou 74. Selon que nous ayons une compétence ou une autre, les règles ne sont pas les mêmes. La compétence du logement n'échappe pas à ce principe. Ainsi la situation du logement à assez Martin singulière entre identité spécialité législative. La compétence du logement est une compétence de la collectivité alors que le social relève du droit commun national. Depuis plus de 10 ans suite à un transfert de compétences en avril 2012. La collectivité voué à fixer les règles applicables dans les Dom. Dans les matières suivantes. Urbanisme de la construction de l'habitation et du logement. Nous ne disposons donc plus de ce fait des dispositifs d'aide à la Pierre. De la LBU. Pas de dispositif financier au titre de la RH ni de la pomme. Au-delà de la complexité engendrée par ce transfert massif c'est Martin pâtit de manque d'accompagnement de l'État non sollicités, je dois l'avouer. De transfert des charges non compensées et le cyclone dévastateur peu après. Il en est juste pour le territoire un déficit de logement social, mais aussi le logement intermédiaire. Si la collectivité a du mal à s'approprier la compétence logement au sens large. Je reste convaincu que nous devons refonder les cadres d'action de la politique du logement à Martin avec l'aide de l'État, par le biais de conventionnement sous des programmes spécifiques. Aussi, nous devons continuer à avancer sur 3 convention tripartite. La convention comme État Action logement que nous devons signer je l'espère rapidement la convention comme État Anna la convention comme État ANRU. Nous aurons dans ces 3 cas besoin de l'ingénierie administrative de l'État.-- Et mais aussi de votre appui, Monsieur le Ministre pour pouvoir avancer. La participation des employeurs à l'effort de construction. P E. Appelé également dispositif de hein du 1% logement est également une piste de travail pour le territoire de Saint-Martin. Il en aurait actuellement 8 entreprises éligibles sur le territoire dans une entreprise de plus de 250 salariés, ce qui équivaudrait hein 2022 à une recette de 88.000 euros. La participation de l'employeur pourrait s'effectuer via un versement un organisme collecteur agréé généralement appelés organismes du 1% patronal.-- En comptant le plan d'investissement volontaire d'Action Logement pourrait nous permettent de récupérer à Saint-Martin entre 2 millions, 5 et 3 millions par an sur les 5 prochaines années. Il est en effet impératif que la collectivité de Saint-Martin puissent bénéficier du reliquat de 400 millions du plan d'investissement 2019 2020 qui je l'espère, Monsieur le Ministre, sera prolongée en 2023 2024 nous attendons d'ailleurs à être rassurés sur ce point. En fait, il pourrait être possible de bénéficier, à l'instar de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon également régies par l'article 74 de crédit, l'État au titre de la rénovation de l'habitat insalubre. En insistant sur l'angle de la politique publique de compétences étatiques. La problématique du logement insalubre. À Saint-Martin justifierait cet effort supplémentaire de l'État. Monsieur le Ministre ainsi présenter les actions prioritaires ou c'est Martin qui pourrait sensiblement amélioré la solution du logement des Saint Martinois je vous remercie. Merci cher collègue. Monsieur le Ministre. Ministre. La sénatrice Petrus. Je vois que vous copiner avec le président Artano qui a à peu près les mêmes problèmes à à Saint Pierre et Miquelon. Hein, et on va essayer d'y travailler. Je dois rencontrer prochainement le président Mussington ici à Paris pour évoquer tout cela. Vous avez raison, il y a des règles à changé hein et c'est cela dont nous avons parlé dans la suite du 7 septembre et du. Appel de Fort-de-France. Ça ne va pas vous avez pas accès à un certain nombre de sujets allant rue à la a notamment vous avez pas accès. Auprès d'Action Logement. À 0 45. Mais vous le président Mussington et décidé. À à souhaiter que ces entreprises puissent cotiser hein puissent cotiser. C'est d'ailleurs pas un problème de recettes. C'est un problème d'avoir accès à l'ensemble des prestations d'Action Logement. Donc, nous y travaillons l'Lana l'ANRU Action Logement. Et. C'est le sujet du débat que j'aurai avec chacun, je le répète des préjugés voit le président l'aider à se à Saint Barthélémy. Je vois le président Mussington chez vous je vais demain, je leur ai dit j'ai en fait trois dans la dans les 15 jours qui viennent travailler sur ces sujets, je voudrais en profiter. Madame la sénatrice, pour dire au président Mussington. Comme je l'ai dit à. Saint-Pierre-et-Miquelon comme je le dis à Saint-Barth. Il faut qu'il me donne des terrains. Si tu veux. Sinon on n'arrivera pas à loger les fonctionnaires.

Un bail emphytéotique. Il les donne à des cibles des agents des promoteurs immobiliers, que j'ai trouvé qu'ils sont capables de rendre. L'ensemble des constructions au bout de 50 ans, la collectivité si des terrains qui sont propriété des collectivités locales, ça coûte rien à personne. Il y a des investisseurs qui sont prêts à faire du logement

part de ne pas remercier la Commission d'avoir autorisé cet échange.-- Né du ciel. Je viens juste écouter ce qu'il a à faire.-- Je viens écouter ce qu'il a à faire et si c'est pas vous qui me le dites, alors on va écouter les administrations vous faire de l'administration administrante. Ça va être sympa donc.-- Merci président. De cette occasion d'échanges c'est fondamental. Derrière. Il nous faut modifier. On a commencé y'travailler dans l'administration, on a commencé il travailler avec d'autres ministères. Il nous faut modifier cette approche. Nous ne réussirons pas tout de suite.-- Ce sujet du logement. Et Lurel va le redire, il est vous l'avez tous dit il est au coeur.-- De l'avis des habitants une est au coeur de ce qui sont. Et ça doit être différencié. Non je pense qu'on va y arriver. Dans le cas de tout ce qu'on s'est dit. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'organisation. C'est un problème de volonté, d'organisation. LBU, enfin on l'a consommé. consommé. Pas si on va y arriver en 2022 mai sur 20 21 ans la on c'est pas un sujet d'argent il y en a on en prend, c'est vraiment un sujet d'organisation de volonté différenciation de travailler ensemble de règles de normes. C'est ça qui compte.-- Moi j'y suis prêt, j'arriverai pas sans vous.-- J'y arriverai pas sans les collectivités locales. J'y arriverai pas sans les constructeurs.-- Je crois profondément, profondément.-- Que cette décision. Que j'ai prise au moment de préparer cette soirée.-- De quitter le plan. Pour aller à un objectif logement telle qu'on la décrit. Cosigné par tout le monde.-- Avec certes un. Chapeau général mais après territorialisée.-- Pour ah nous permettent d'avancer. Personne n'est jamais sûr de réussir, mais en tout cas ce que je voudrais c'est que.-- On soit convaincu qu'on a plus de chances de réussir si on est ensemble que si juste on fait. Des grandes déclarations, y compris, ça vaut pour l'état hein, ça vaut pour l'État bien sûr. Voilà c'est ce que j'ai, j'essaie de faire et je voudrais conclut en disant.-- Merci, merci de me pousser, de pousser les administrations de pousser l'État. À bouger tout seul on reste cool hein. Voilà donc merci à.-- Merci, monsieur le Ministre. La parole. Donc pour conclure est à Monsieur Victorin Lurel au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Monsieur le président de la délégation. J'ai un collègue. J'avoue que je suis bien gêné. C'est bien la première fois que j'ai à conclure un débat et je sais pas quoi vous dire. Et quoi vous rapporter. J'avoue que je suis assez. C'est vrai que j'ai eu du plaisir à réécouter puisqu'il avait des phrases de poésie et ça nous intéressait. Mais. Je suis un vieux parlementaire et j'avoue que je suis assez étonné par la prestation de notre ministre. Absolument. Et j'avais préparé un très beau discours. Je crois que je vais le laisser. Parce que c'est pas la peine de répéter ce que vous savez ce que nous savons tous et au moins vous dire 2 ou 3 petites choses, la première chose. Je demanderai à mon ministre à notre ministre. Vous êtes ici au Sénat. D'éviter. Quelques sorties. Qui peuvent si elles avaient été prononcés à l'Assemblée nationale ou dans d'autres, en fait qui pourrait faire débat. Parler de la pression migratoire en Guyane des Syriens des Kurdes. Et des. Il y avait une autre nationalité au prix de la cathédrale. J'ai une conversation et la pratique. Mais dans un centre un temple républicain comme celui-là, évitons ces approximations. Ça c'est une première chose, il faut régler les problèmes, on les connaît depuis de très longues années, moi je suis restée 15 à l'Assemblée nationale. Six ans ici ça fait une vingtaine d'années, on connaît les problèmes. Monsieur le Ministre, vous êtes là depuis 7 mois. Vous avez eu un prédécesseur, qui a eu lui-même des policiers. Et moi aussi j'ai occupé votre en fonction. On sait vous n'arrivez pas pour découvrir les problèmes que vous. À vous écouter monsieur le Ministre, vous êtes d'accord sur tout. Vous aviez par exemple. Satisfaire aux demandes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Depuis fort longtemps, on connaît aux alliés de nous faire.

On n'a pas réglé le problème. Vous voyez, vous avez. Ne. Non, non vous ne pouvez pas Monsieur le Ministre. La seule instance non non on a choisi d'ignorer. Cette instance là. Tous les parlementaires ici à l'Assemblée nationale. Tous les acteurs et beaucoup de maires des autres ont signé. Non, vous demandez à arrêter un contentieux. Je suis d'accord mais faites-le. Oui. Choisissez aussi des représentants pour que nous puissions défendre nous c'est pas le cas. À vous écouter, nous allons. Faire intervenir. Comme maintenant le multiples acteurs. Monsieur le Ministre, Georges, vous dire que vous n'arrivez jamais à régler ce problème, parce que vous n'êtes pas compétent surtout en permettez-moi de vous dire et d'être un peu estomaquée parce que vous dites. oui mais l'État n'est né. Pas seule responsable, bien sûr on a jamais dit ça. Mais la politique du logement et notamment de l'audience. Ça reste une politique de l'État elle est verticale, elle est centralisé et Catherine qu'on qu'on ne l'a dit excellemment. Elle est centralisé. Alors moi j'ose vous dire dans une synthèse. Après 77 recommandations. Un excellent travail fait par la délégation que nous vaudra peut-être pas suffisamment lu puisque vous n'avez retenu jusqu'ici aucune mesure proposée. Moi je ne sais pas qu'est-ce qui est entrée en application mais avant vous, il y avait un ministre il y a une continuité de l'action de l'État, vous avez pris un relais vous n'inventez pas tout. Moi, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous avez monté tous vous Découvrez tout. Vous allez tout régler je découvre, là je suis peut être pas le seul que le plan 3 après un plan eux qui a été un échec. J'étais à l'origine de ça pour a pris la suite. Tous les ministres ont, ont pris la suite le plan de n'a pas été exécutés, les comités de pilotage et vous êtes aussi coresponsable n'ont pas été. 0 échec total parce que ils n'. Maintenant il y aura non plus hein. L'homme droit mais un objectif logement outre-mer on nous avons faire un empilement de choses que nous savons, il n'y a pas donc finalement d'orientation. Je vous propose ce que tous les collègues nous ont dit ce que Catherine qu'on nous a dit faites une révolution systémique. Comment voulez-vous en traitant les gens un adulte que vous à l'époque, c'était 243 millions ACP vous avez 179 millions, vous avez dit qu'il y a pas d'ingénierie et ben vous baisser de 3 millions aujourd'hui, les crédits consacrés à l'ingénierie. je pense plutôt que tout ça c'est une manière de se défausser de dire je suis pas seule responsable, je vous propose, nous vous proposons un adulte, un responsable avec le sens donc des responsabilités, de décentraliser de délégués de faire la dévolution des crédits de la LBU. On l'avait pris de ministère du Logement, vous le, je sais bien ça posera problème le ministère alors créer un ministère de la mer et des Outre-mer mettez des préfectures maritimes ça donnera de la mission de l'activité la des JO même n'a pas les moyens pour s'occuper en temps réel de nos problèmes. Monsieur le ministre vous demande que l'objectif logement soit soumis aux parlementaires soient soumis à notre délégation pour que on, on vous donne quelques. Quelque ambition et puis de le faire très vite, vous avez voté un budget, vous l'avez aux côtés, hé bien on attend beaucoup plus que ça. Monsieur le Ministre, chers amis, je me permets de le dire, il est temps d'agir. Alors il faut se réveiller. Merci cher collègue. Merci. Merci pour ce débat. Je vais lever là c'est la séance. Mes chers collègues. La prochaine séance jeudi 12 janvier, 2023 10h 30 pour les questions orales. La séance est levée.